Mes chers collègues, lors de sa réunion du 28 janvier dernier, la conférence des présidents a donné son accord pour que le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, inscrit à l'ordre du jour du mardi 3 mars, fasse l'objet de la procédure de législation en commission partielle. Réuni le 18 février, le bureau de la commission spéciale a établi une liste de dix articles pouvant faire l'objet d'un examen selon cette procédure. Elle a été communiquée aux groupes politiques, qui n'ont pas formulé d'opposition. Les articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49 feront ainsi l'objet de la procédure de législation en commission. le délai limite pour le dépôt des amendements de commission au lundi 24 février à douze heures, la date de réunion de la commission pour le rapport et le texte au mercredi 26 février à seize le délai limite pour le dépôt des amendements de séance portant sur les articles du texte non concernés par la procédure de législation en commission au lundi 2 mars à douze heures, le délai limite de demande de retour à la procédure normale pour les articles faisant l'objet de la procédure de législation en commission au vendredi 28 février à dix-sept heures. Y a-t-il des observations ?

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

celui de faire comprendre que cette profession avait une attente forte, une attente que nous pourrions résumer par un mot : la reconnaissance. Les États généraux de l'agriculture qui se sont tenus peu après ont amplifié cet espoir,

Qu'allez-vous proposer sur les risques et les aléas ? Allez-vous défendre l'assurance récolte, le stockage de l'eau, l'irrigation, les progrès s'agissant des semences, alors même que le Conseil d'État, par exemple, vient de les classer OGM ? Monsieur le ministre, je suis conscient que votre tâche est difficile. À mon modeste niveau, si j'étais à votre place, je ne me poserais qu'une seule question

Premièrement, soutenez que la production agricole française est diversifiée et arrêtez d'opposer les agriculteurs entre eux. Surtout, cessez de dire que vous voulez changer de modèle. Très bien ! Notre modèle est fort quand il est fort à l'export et quand il est défendu par son ministre. Le savoir-faire français rayonne, il se vend. Profitons-en ! N'oublions jamais que 25 % du revenu des agriculteurs dépend de la capacité exportatrice de la France. Notre modèle agricole différencié est fort, en France, quand il est respecté, quand on allie proximité, circuits courts, restauration hors foyer, qualité des AOP, du bio, mais aussi du conventionnel et du traditionnel. Deuxièmement, il faut lutter contre la suprématie des quatre centrales d'achat.

Si nous ne voulons pas voir ce que le progrès peut nous apporter, nous sombrerons dans l'obscurantisme. Les craintes des consommateurs peuvent trouver leur réponse dans la recherche et dans l'innovation.

Ne les combattez pas ! Au contraire, faites-en une force, avec une vision et un projet, et, vous verrez, ils vous surprendront.

de travailler pour les pêcheurs, pour les conchyliculteurs, pour l'ensemble du monde agricole, pour les forestiers, pour les entreprises agroalimentaires et pour l'agroalimentaire. Voilà l'enjeu de la politique menée par le Gouvernement ! Il s'agit d'abord d'écouter, de comprendre et d'accompagner les agriculteurs, parce que ce sont ceux qui font l'agriculture, ceux qui travaillent dans l'agriculture, ceux qui travaillent pour l'agriculture qui sont les plus à même de parler de l'agriculture, même s'il n'est pas forcément utile d'être agriculteur pour comprendre la dynamique agricole et pour travailler

aux instructions données par la garde des sceaux pour lutter contre toutes les intrusions, contre le dénigrement, contre toutes les attaques dont font l'objet les agriculteurs. Le premier engagement, c'est évidemment celui de la transition agroécologique. Nous ne voulons pas changer de modèle,

on ne fait pas muter l'agriculture au rythme des tweets, on fait muter l'agriculture au rythme des saisons, au rythme des pratiques culturales. Dans cet hémicycle, comme à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas tous les mêmes positions.

il faut que celle-ci s'appuie sur un triptyque : la compétitivité, la recherche et la transition agroécologique. Sans compétitivité, sans création de valeur, sans création de richesses, l'agriculture sera par terre. Mais cette agriculture ne pourra se faire que si l'enseignement supérieur et la recherche

aux commissions des affaires européennes et des affaires économiques, a fait des propositions au Gouvernement et à la Commission européenne sur le budget et les règles de la prochaine PAC. Le cadre financier pluriannuel de la nouvelle Commission européenne va se traduire par des diminutions budgétaires très sensibles pour les aides directes : de l'ordre de 15 % pour le premier pilier et de 25 % pour le développement territorial, qui comprend les aides à l'installation, à la conversion au bio et l'accompagnement des territoires ruraux. Par ailleurs, la nouvelle gouvernance de la PAC nécessitera que les États membres présentent à la Commission leur plan stratégique. Ma question est simple, sur quels principes ou dispositifs allez-vous construire le plan stratégique agricole de la France afin d'améliorer le niveau et la stabilité du revenu des agriculteurs et de renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires, de mettre en oeuvre les 40 % des budgets du P1 et du P2 qui devront être consacrés aux problématiques environnementales et climatiques- je pense notamment au de Mme von der Leyen -et pour soutenir le niveau du marché du bio, qui s'accroît en volume mais qui baissera inéluctablement en valeur, donc en termes de revenus pour les producteurs

Monsieur le ministre, avec l'ensemble des viticulteurs de mon département du Gers, je souhaite que vous preniez la mesure des difficultés auxquelles ces viticulteurs sont confrontés malgré les efforts considérables qu'ils font pour répondre aux marchés nationaux comme lointains- je pense notamment aux labels HVE 3 et aux conversions au bio. Ne laissons pas cette filière, qui est l'un des fleurons de notre agriculture et de notre commerce extérieur, sans accompagnement immédiat. Réagissons sans attendre, en activant peut-être la réserve de crise européenne.

Parmi celles-ci, je souhaite évoquer la question de l'emploi agricole. Aujourd'hui, devenir agriculteur n'est plus nécessairement une destinée. En outre, dans une France désormais largement urbaine, la vocation aux métiers agricoles n'est plus évidente, et ce d'autant moins qu'ils véhiculent une image de pénibilité et de faibles rémunérations, liée aussi à un agribashing dévastateur. Notre agriculture ne fait pas rêver nos jeunes, sans parler des suicides qui l'endeuillent chaque jour. Aussi, si nous voulons porter une ambition forte pour notre agriculture, n'oublions pas l'essentiel : pourvoir le secteur en main-d'oeuvre. d'une main-d'oeuvre adaptée aux nouveaux enjeux, en particulier ceux qui sont liés à l'innovation, à l'agroécologie, à la polyactivité, à l'évolution du cadre juridique de l'exploitation, à l'essor numérique ou simplement à la conduite d'engins agricoles. Quel soutien public faut-il aujourd'hui pour que les exploitants ne se retrouvent pas confrontés à une pénurie de main-d'oeuvre ? Près de 70 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues. Dans ces conditions, il faut nous interroger sur nos politiques publiques. Je mesure régulièrement cette faiblesse sur le terrain alors que la question du chômage est particulièrement prégnante au coeur de nos territoires ruraux, les agriculteurs doivent de plus en plus souvent recourir à de la main-d'oeuvre étrangère organisée, avec tout ce qu'elle suppose de précarité pour les salariés étrangers. C'est désolant Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais connaître les actions concrètes que pourrait prendre le Gouvernement pour réconcilier au plus vite l'offre et la demande d'emploi dans l'agriculture et redorer son image. L'agriculture a besoin d'agriculteurs- de bras, oserai-je dire. J'attends vos réponses sur le volet de l'emploi, essentiel à la survie de l'agriculture française. monsieur le ministre,

Force est de constater que les résultats sont pour l'instant insuffisants- vous l'avez d'ailleurs fait remarquer -, en particulier dans certaines filières. J'aimerais ici aborder le cas de la filière bovine. La mise en oeuvre d'une mesure phare de la loi Égalim, à savoir l'inversion de la construction du prix, se heurte, au sein de l'interprofession, au blocage des industriels et de la distribution. L'objectif, qui était de sanctuariser la prise en compte des coûts de production et de ne plus partir de la marge que souhaitent dégager les transformateurs et les distributeurs, n'est manifestement pas atteint. Certaines organisations représentant les industriels et la distribution utilisent leur droit de veto afin de bloquer les méthodes de calcul ainsi que la prise en compte des coûts de production. Alors qu'est confié aux interprofessions le rôle de rédiger des plans de filière, ces méthodes empêchent toute perspective d'amélioration du revenu des producteurs, à l'instar de nombreuses filières. Aucune contrainte n'est prévue dans la loi, et l'État ne s'est pas doté de véritables moyens de pression. Monsieur le ministre, quels sont les leviers d'action du Gouvernement pour motiver les interprofessions à mieux s'organiser au profit du producteur ? Comment peut-on remédier à ces blocages pour pouvoir enfin évaluer le potentiel de cette loi Égalim ?

Les années qui viennent ne feront pas exception. Alors que les négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel se poursuivent, avec des points de vue bien différents, et que la réforme de la politique agricole commune est également en discussion, l'agriculture constitue un point central où la France doit occuper une place de chef de file. La Commission européenne a présenté en décembre dernier son pacte vert européen, ambition se mêle à réalisation. Nous devrions donc connaître, dès mars 2020, la stratégie « de la ferme à la fourchette », qui sera révélée au même moment que celle pour la biodiversité, ou encore celle sur l'industrie européenne. Autant de sujets que l'Union européenne va devoir gérer en même temps, tout comme le verdissement de la PAC, la neutralité carbone, notre indépendance et notre sécurité alimentaires, l'aide aux agriculteurs, la lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur agricole et la transition énergétique, pour ne citer que ces défis dont la liste est bien plus longue. En somme, les questions agricoles sont au coeur des évolutions européennes. Elles sont à la croisée des chemins de bien des stratégies que l'Union européenne souhaite mettre en place. La question agricole est notre futur commun.

la réforme de la PAC, son financement et les exigences principales du nouveau pacte vert européen

pour la transition écologique reposait sur la transition agricole au travers d'une logique et d'une action en faveur d'un renforcement significatif de la qualité de nos modèles, tout en préservant notre souveraineté. Cette volonté clairement énoncée a cependant été édulcorée, il me semble, par la perspective d'une mise en application qui doit, en même temps, satisfaire l'ensemble des parties concernées, à l'international comme au niveau européen. Aujourd'hui, nous constatons régulièrement, à la fois, la mise en place de nouvelles contraintes pour nos agriculteurs et la possibilité offerte à des produits ne respectent pas nos conditions de production et ne sont pas soumis au même contrat social de franchir nos frontières. Aussi, cette vision d'ensemble soutenue par le Président de la République ne peut que soulever des inquiétudes. En effet, cela ne signifie-t-il pas une certaine perméabilité à l'idée qu'il faudrait approuver des produits répondant à des normes plus souples

Pourriez-vous également nous garantir qu'aucune nouvelle mesure franco-française ne viendra alourdir un peu plus la situation du monde agricole confronté à des produits qui ne respectent pas le modèle que nous défendons ? comment abordez-vous l'application concrète de l'article 44 que nous avons introduit dans la loi Égalim, qui interdit la commercialisation de denrées alimentaires ne respectant pas la réglementation européenne ?

permettez-moi d'appeler votre attention sur les difficultés structurelles de la filière viande bovine française. Nous ne pouvons pas nous résigner au constat d'un marasme économique sans fin. Nous le savons, les causes de celui-ci sont nombreuses. Elles tiennent en particulier au décalage entre l'offre et la demande de viande de boeuf sur le marché français, à l'absence de stratégie de développement pérenne à l'exportation, au long attentisme de l'interprofession, au du modèle économique des principaux industriels et distributeurs, mais également- je dois le concéder -à l'individualisme de nombreux éleveurs. Une partie de la solution à ces problèmes structurels réside au niveau européen. Nous devons faire en sorte que la future PAC prenne en compte l'exception agricole au regard du droit de la concurrence, sur le modèle du américain de 1922. Fort heureusement, ces dernières années, nos collègues du Parlement européen sont parvenus à faire bouger les lignes à deux reprises : avec l'adoption du règlement Omnibus de 2017, tout d'abord, et celle de la directive d'avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales, ensuite. Pourtant, il nous faut aller encore plus loin en modifiant fondamentalement les dispositions du règlement du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Il conviendrait en quelque sorte de mettre fin à deux verrous d'abord, la faible capacité à agir des organisations de producteurs pour améliorer les prix de vente des producteurs ; ensuite, l'impossibilité pour les autorités françaises d'accroître « en solo » les incitations financières en faveur desdites OP. Mes questions sont claires, monsieur le ministre, j'attends des réponses claires. La parole

lors de la remise des prix d'excellence du concours général agricole au ministère de l'agriculture, il y a un mois, a parlé pour la première fois de l'« exception agricole et agroalimentaire française », au même titre que nous parlons d'exception culturelle.

pour nos vins et spiritueux. Dans ce dossier, un accord est vivement souhaité, afin de préserver les flux, la logistique et les accords de protection de nos IG. Il

La coopération agricole considère que cette ordonnance détricote le statut coopératif, dès lors que celle-ci se trouve banalisée comme un opérateur économique commercial, sans que l'on prenne en compte sa spécificité.

de qualité agronomique médiocre, de primes PAC classiques et de revenus tirés d'une activité photovoltaïque, par exemple. Je pense notamment à un projet, qui est cher

le pays du vin par excellence. C'est notre pays qui bénéficie de la meilleure image dans le monde. C'est pourquoi les nuages qui obscurcissent l'horizon du vin français doivent être dissipés sans attendre. Dans le cas des USA et du Royaume-Uni, nul ne peut le faire à votre place. Cela étant, nous savons tous ce que rapporte la viticulture française en termes d'emploi et d'excédents pour notre balance commerciale. Il faut donc vraiment faire le maximum, monsieur le ministre.

ambassadrice du Canada en France, sur l'Accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, de nombreux échanges ont eu lieu sur l'impact du CETA sur l'agriculture française. À cette occasion, plusieurs de mes collègues ont souligné la souffrance de notre secteur agricole et, plus particulièrement dans le contexte du CETA, de la détresse ressentie par la filière bovine. En effet, celle-ci craint que la ratification du traité ne lui porte un coup considérable, dans un contexte où elle subit déjà une forte pression. Nous avons tous en tête l'hostilité, voire parfois les violences subies par les professionnels du secteur, les normes sans cesse plus exigeantes et les difficultés pour traiter à égalité avec les acteurs de l'agroindustrie, le tout dans un contexte où les attentes des consommateurs sont de plus en plus élevées. Au-delà des enjeux du CETA, les difficultés rencontrées par la filière bovine ne démontrent-elles pas la fragilité de notre modèle ? Comment le Gouvernement se propose-t-il d'agir pour la soutenir ? La loi Égalim constitue un pas dans la bonne direction, mais elle n'est visiblement pas suffisante. La parole

je souhaite vous relayer les préoccupations des agriculteurs et des élus que nous sommes. Les syndicats demandent un moratoire jusqu'à la prochaine période culturale et refusent d'appliquer une réglementation imprécise, avec des appréciations divergentes entre l'administration centrale et les services déconcentrés de l'État, comme ce fut le cas pour les pesticides cupriques. Il aura fallu attendre plusieurs semaines pour que les instructions confirment que l'application de ces pesticides ne sera pas soumise aux distances de sécurité, sauf mention expresse de l'autorisation de mise sur le marché. Par ailleurs, la question du lissage du cuivre n'a toujours pas été réglée. Une instruction, c'est bien ; mais les viticulteurs demandent un texte qui les sécurise juridiquement. Les élus sont, quant à eux, sollicités par certains de leurs administrés pour faire appliquer la loi, alors que les chartes départementales ne sont pas actées. pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ? Les agriculteurs et les nouvelles générations qui s'installent sont de plus en plus sensibilisés aux questions environnementales : ils modifient leurs pratiques culturales et investissent dans du matériel plus performant, mais très coûteux, qui permet de réduire la distance de non-traitement. Or la liste des matériels a été publiée avant la sortie des textes. Elle ne vise que les appareils permettant une réduction de la dérive de 66 %. Quant aux haies comme moyen de réduction de la dérive, elles ne sont pas mentionnées. Il est donc nécessaire de revoir cette liste rapidement. La profession agricole demande une compensation économique et souhaite déclarer les zones non traitées en surface d'intérêt écologique (SIE), en jachères, en prairies ou en mesures agroenvironnementales. Enfin, il est difficile d'imposer à nos agriculteurs des mesures restrictives et de laisser entrer sur le marché français des produits alimentaires traités avec des substances interdites sur notre sol, en totale contradiction avec l'esprit de la loi Égalim- cela a été dit précédemment. Le dialogue, la concertation et la voie de la raison doivent être de mise. Il y va de la cohésion sociale et du bien vivre ensemble dans nos territoires. Monsieur le ministre, nous attendons des réponses claires et précises, car il y a trop d'incertitudes sur les modalités de mise en oeuvre et d'insécurité juridique

j'ai rencontré l'ensemble des organisations professionnelles agricoles- le Président de la République aussi -afin de leur expliquer clairement la situation. D'abord, je vais vous dire une chose : si nous en sommes là, c'est parce que la France a été condamnée par le Conseil d'État. Il faut toujours le rappeler, car, moi, je veux bien tout

la commission des finances du Sénat a donné son accord à la publication d'un rapport sur les financements publics accordés à l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est désormais une activité majeure dont l'importance va croissant. Elle représente une opportunité économique pour les agriculteurs et répond par ailleurs à des attentes sociétales très fortes. Les pouvoirs publics lui ont fixé des objectifs contenus dans le programme Ambition bio 2022 ils se résument en deux chiffres : 15 % de la surface agricole utile (SAU) devra être convertie en bio en 2022 et la part du bio dans la restauration collective devra atteindre 20 %. Or, si l'on se réfère à l'évolution de la conversion des terres, ce n'est pas avant 2026 que cet objectif de 15 % de la SAU en bio sera atteint. Dans le même temps, la France importe 30 % des produits bio qu'elle consomme. Le moment est donc venu de clarifier un certain nombre de points et de lever quelques freins. la question des moyens budgétaires de soutien aux agriculteurs bio est à remettre à plat. Aujourd'hui, tout ou presque passe par l'Europe, les régions, voire les agences de l'eau : ces aides sont dispersées et mettent trop de temps à être versées aux bénéficiaires. En second lieu, il faut garantir la sincérité des produits bio entrant en France. La confiance du consommateur, donc la fiabilité et la pérennité de la filière, passe par un renforcement des contrôles de la DGCCRF, dont les moyens doivent être adaptés.

La situation de l'ITAB, l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologiques, est fragile. Or son rôle est stratégique en matière de recherche et de développement. Quels moyens seront mis en place afin d'accompagner la recherche ?

subjectif et comporte une dizaine de comme l'on dit aujourd'hui. Je suis au regret de vous le dire, d'autant que je n'aime pas polémiquer et que je connais votre exigence intellectuelle. Ce rapport m'a beaucoup choqué

La délégation en avait fait état dans un rapport très étoffé en 2017. Selon les informations transmises voilà trois ans par votre ministère à la délégation, seuls 31 % des agriculteurs et des agricultrices totalisaient une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres, soit 37,5 années. Avec Avec la mise en place d'un système universel à points et l'obligation d'avoir accompli une carrière complète, ne va-t-on pas aggraver encore la faiblesse des retraites agricoles, singulièrement celles des agricultrices ? Nous ne pouvons en effet ignorer que les agricultrices embrassent cette profession souvent plus tardivement que les hommes. Un autre sujet d'importance est celui de la liquidation des pensions. Lorsque nos collègues de la délégation ont publié leur rapport sur les agricultrices en juillet 2017, une réforme venait d'entrer en vigueur : la liquidation unique des retraites des régimes alignés. Il s'agissait alors de simplifier la liquidation des pensions de retraite pour les polypensionnés et de permettre aux assurés des régimes alignés de liquider l'ensemble de leur retraite de base en s'adressant au dernier régime d'affiliation pour obtenir un paiement mensuel unique de leur pension. Dans son rapport, la délégation avait toutefois exprimé la crainte que cette réforme ne se traduise par une baisse des retraites pour certaines agricultrices, relativement nombreuses parmi les personnes polypensionnées. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ? Pouvez-vous également nous indiquer ce qu'il adviendra de cette liquidation unique avec le système à points ? La parole Monsieur le ministre,

85 % du SMIC, ce n'est pas une grande revendication. Je m'adresse à nos deux collègues communistes présents dans l'hémicycle : voilà deux ans,

sans attendre la fin des discussions sur les retraites. La occasion de mettre à l'honneur ce beau métier que celui de nourrir nos concitoyens et qui demande cinquante à soixante-dix heures de travail par semaine, je voudrais focaliser mon intervention sur l'agribashing, évoqué par Laurent Duplomb et certains de nos collègues. Cette attaque en règle de notre agriculture et de la ruralité prend la forme de harcèlements permanents envers nos agriculteurs, que ce soit de la part de mouvements extrémistes extrémistes végans ou des « faucheurs volontaires ». Ceux-ci mènent des campagnes d'intimidation inacceptables, sous forme d'actions violentes à l'encontre de certaines professions, dont les bouchers, mais aussi les agriculteurs, qu'ils soient éleveurs ou céréaliers. Ces six derniers mois, ce ne sont pas moins de soixante interventions malveillantes dans les fermes qui ont été constatées. Parallèlement, les fermiers se voient régulièrement cambriolés. On leur vole du fioul, des capteurs GPS, encore le week-end dernier près de chez moi, dans le département de l'Aisne, du matériel, des véhicules agricoles ou encore du bétail. Récemment, dans la Marne, un éleveur, parce que déjà cambriolé plus de quarante fois depuis 2015, a grièvement blessé au fusil le dernier cambrioleur. Le contexte particulièrement anxiogène. C'est en partie une des raisons, en plus de celles qui ont été évoquées par tous mes collègues, pour lesquelles les exploitants et les salariés agricoles ont un risque plus élevé de décès par suicide que l'ensemble de la population- un par jour, je le rappelle, et ce depuis plusieurs années

et une action en faveur d'un renforcement significatif de la qualité de nos modèles tout en préservant notre environnement. Néanmoins, il ne faut pas que cette évolution se traduise par un environnement économique dégradé pour nos agriculteurs, qui subissent déjà trop de changements et qui ne peuvent assumer sans cesse de nouveaux ajustements.

des zones de non-traitement : pouvez-vous nous garantir que leur mise en place ne se traduira pas par de nouvelles charges ? Le cas échéant, quelles mesures concrètes de compensation financière des éventuels surcoûts prévoyez-vous ? Pouvons-nous compter sur des mesures d'accompagnement, tel qu'un plan global d'investissement dans du matériel adéquat, dans la durée et pour toutes les filières ? En second lieu, la réglementation des zones de non-traitement au 1 janvier 2020 s'analyse indubitablement comme un mauvais signal envers les agriculteurs, qui doivent encore et toujours s'adapter

Aussi, pouvez-vous nous garantir que l'implantation de ces zones de non-traitement se fera sans consommation supplémentaire de foncier agricole et que, le cas échéant, les aménageurs incluront dans l'emprise de chaque projet l'implantation de telles zones ? Monsieur le ministre,

Monsieur le ministre, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous voulez améliorer le quotidien de nos agriculteurs. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux ! Or les comptes ne sont pas bons. En décembre 2019, les prix à la production de l'ensemble des produits agricoles étaient en baisse de 0,4 alors que les prix à la consommation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées augmentaient de 2,1 %. De façon plus générale, la faiblesse des revenus agricoles s'observe dans bon nombre de filières- je n'y reviens pas. À ce propos, la commission des comptes de l'agriculture de la Nation a publié, le 10 janvier dernier, les résultats des exploitations agricoles : le résultat net La loi Égalim ne rééquilibre pas les relations commerciales- force est de le constater. Cette loi laisse même un goût amer aux paysans et elle ne donne pas de perspectives en termes de prix.

que cette loi n'est pas la solution et que nous ne pouvons la laisser en l'état. Monsieur le ministre, ma question est simple : quand le Gouvernement compte-t-il enfin se mettre au travail pour redonner de la dignité à une profession toujours plus précaire ? Les agriculteurs de notre pays attendent des réponses, à l'heure où s'ouvre le salon de l'agriculture, censé promouvoir notre agriculture et le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes qui ont une mission d'intérêt public : nourrir l'ensemble de nos concitoyens. est à M. le ministre. Madame la sénatrice, soyons fiers de notre agriculture, soyons fiers de notre alimentation, soyons fiers de nos agriculteurs. Arrêtons de toujours parler négativement de l'agriculture et des agriculteurs. Le salon de l'agriculture va s'ouvrir. Il va être une formidable vitrine.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans deux jours, le salon international de l'agriculture ouvrira ses portes, et, comme chaque année, les Français seront au rendez-vous. Mais cet engouement ne doit pas masquer la réalité du quotidien des agriculteurs français ; c'est pourquoi les élus du groupe Les Républicains ont souhaité l'inscription d'un débat sur l'action du Gouvernement dans ce secteur.

à elle seule, notre agriculture représente près de 17 % de la production européenne. Elle reste une force exportatrice qui pèse positivement dans la balance commerciale de notre pays. Nous sommes une puissance agricole de premier plan, fruit d'une longue tradition d'excellence, de savoir-faire reconnus dans le monde entier, et près d'un quart de nos exploitations agricoles produisent sous des labels d'identification de la qualité et de l'origine. Notre agriculture est un acteur de la transition énergétique. Elle est respectueuse de l'environnement, elle est même un acteur majeur de sa préservation. Elle répond aux enjeux d'une économie toujours plus circulaire et plus durable. Pour la troisième année consécutive, l'hebdomadaire britannique classe

Leurs revenus subissent une diminution dramatique, malgré les promesses de la loi Égalim. On demande toujours plus à nos agriculteurs, qui affrontent la concurrence déloyale des produits importés. Enfin, la renationalisation annoncée de la PAC soulève des inquiétudes. Or, malgré les sacrifices consentis par la profession, la méfiance de la population envers les agriculteurs est de plus en plus visible. Je vous le demande : quelle est quelle est cette société dans laquelle les données scientifiques reculent devant l'hystérie collective ? Les actions violentes et les agressions d'exploitants doivent nous alerter. Le Gouvernement doit cesser d'alimenter l'agribashing. Or il ne montre pas l'exemple. J'en veux pour preuve vos décisions récentes quant aux zones de non-traitement, dont il a été question au cours du débat. Parce qu'il s'agit d'un secteur stratégique, le Sénat, et particulièrement sa majorité, a toujours eu à coeur de défendre l'agriculture dans ses travaux et de faire des propositions concrètes pour tenter de redresser la barre. Malheureusement, le Gouvernement n'y est pas très réceptif. Un exemple parmi d'autres les travaux de suivi de la loi Égalim ont montré que, avec l'encadrement des promotions, de nombreuses PME et ETI de l'agroalimentaire, particulièrement dans le secteur des produits saisonniers, se trouvent en difficulté. C'est pourquoi une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité du Sénat le 15 janvier dernier, pour contrer ces effets pervers de la loi et, ainsi, sauvegarder l'activité dans les territoires ruraux. Quelle ne fut pas notre surprise de constater dans le projet de loi ASAP, à l'article 44, une prolongation de l'expérimentation de l'encadrement des promotions Lors de la discussion de la proposition de loi, vous nous avez demandé d'attendre la fin de l'expérimentation pour en tirer tous les enseignements. Or, sans aucune évaluation, vous demandez aujourd'hui au Parlement de prolonger un dispositif qui fragilise nos territoires. Ce mépris des travaux du Parlement est malheureusement une marque de fabrique de la majorité présidentielle et de ce gouvernement. Et, dans ce cas, c'est l'agriculture et le secteur agroalimentaire qui en subissent les conséquences. Dernièrement, nous vous avons adressé des propositions sur des sujets précis. En voici deux exemples. deux exemples. Avec notre collègue Yannick Botrel, je viens de déposer un rapport sur l'agriculture biologique, dans lequel nous recommandons de mettre en cohérence les objectifs de conversion des exploitations avec la programmation financière. Les crédits diminuent, alors que la demande de produits bio est en hausse en France, et nous nous voyons forcés d'importer 30 % des produits consommés. Dans son rapport

ou encore de lutter contre la concurrence déloyale des importations ne respectant pas les normes imposées aux agriculteurs français. Monsieur le ministre, nous éprouvons semble-t-il les mêmes inquiétudes et nous dressons les mêmes constats. Joignez la parole aux actes et saisissez-vous des propositions concrètes que formule le Sénat. L'agriculture française et les agriculteurs sont face à des défis majeurs nous devons collectivement, et particulièrement votre ministère, être à leurs côtés et pas seulement sous l'oeil des caméras au salon de l'agriculture ! Nous en

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de nombreux travaux ont été menés par le Sénat ces derniers mois sur le thème de la politique spatiale : notre commission des affaires européennes a publié, l'été dernier, un rapport d'information sur la politique spatiale de l'Union ; un groupe conjoint à la commission des affaires économiques et à la commission des affaires étrangères a produit un rapport invitant à restaurer l'ambition européenne dans le domaine des lanceurs l'Opecst a également publié plusieurs notes de grande valeur sur le sujet, notamment sur les satellites et les lanceurs. De fait, l'année 2019 a représenté un cap pour l'Europe spatiale, puisque Ariane a brillamment passé la barre des 250 lancements, ans après sa mise en service. La fin de l'année a été marquée par le succès de la conférence interministérielle de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, à Séville ; j'y reviendrai. Si la commission des affaires européennes a souhaité que soit organisé aujourd'hui un débat sur la politique spatiale européenne, ce n'est pas seulement pour se réjouir de ces succès, mais aussi pour que nous portions ensemble un regard prospectif sur les défis à venir. Ceux-ci sont nombreux, et, nous en sommes convaincus, ce n'est qu'à l'échelon européen que nous pourrons y apporter une réponse. Les outils et les données fournis par l'activité spatiale sont indispensables pour affronter des enjeux qui ne peuvent eux-mêmes être envisagés et traités qu'au niveau européen. Je pense, par exemple, au changement climatique : sur cinquante variables essentielles pour mesurer le changement climatique, vingt-six ne peuvent être observées ou mesurées que depuis l'espace. Les satellites sont aussi seuls capables de mesurer de nombreux paramètres concernant les océans, où il peut être difficile de recueillir des informations : acidification des eaux, évolution des glaces de mer, prolifération des algues ou modifications du trait de côte, autant de variables dont l'analyse est un enjeu essentiel pour la planète. Le spatial nous donne alors les moyens d'améliorer la prise de décision politique. Un autre exemple est l'internet par satellite, qui peut contribuer à la réduction de la fracture numérique. Le spatial offre dans ce domaine des moyens techniques pour mettre en oeuvre nos décisions politiques. Le spatial et les applications qui en sont issues touchent aussi des domaines plus sensibles. Une politique spatiale ambitieuse est donc indispensable pour assurer l'autonomie stratégique et la sécurité de l'Europe, dont l'indépendance même est, à terme, en jeu. Il ne s'agit pas seulement de la militarisation de l'espace, mais aussi d'assurer, par exemple, la continuité de nos moyens de communication. il faut saluer le programme initié par la Commission européenne, GovSatCom, qui devrait être en mesure de fournir, dès 2020, des services sécurisés de communication par satellite aux pays, organismes et opérateurs d'importance vitale de l'Union. Au-delà de ces programmes ciblés, il est indispensable que l'Union européenne demeure un acteur de premier plan de toute la chaîne de valeur du secteur spatial. Des signaux positifs ont été envoyés ces derniers mois par les États comme par les instances européennes, marquant une véritable prise de conscience de l'importance du secteur spatial. Nous pouvons saluer, au niveau de la Commission européenne, la mise en place d'un règlement unique pour l'ensemble des activités spatiales de l'Union et la création d'une nouvelle direction générale- Defis -, spécifiquement dédiée aux industries spatiales et de défense, placée sous la houlette du commissaire français, Thierry Breton. Néanmoins, trois points méritent notre vigilance. Le premier est celui de la gouvernance. Nous avons tous en mémoire l'interruption de service de Galileo l'été dernier, causée par des problèmes de coordination entre les différentes parties prenantes. Il est donc nécessaire de rationaliser cette gouvernance, notamment en précisant le rôle de la future Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, l'Euspa. Les prochaines négociations entre la Commission et l'ESA, agence interétatique dont le périmètre ne recouvre pas celui de l'Union, s'annoncent difficiles sur ce point, encore plus depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le deuxième point est celui du financement. Les États-Unis, leader historique, consacrent chaque année plus de 40 milliards d'euros au secteur spatial, la Chine, qui ne cache plus ses ambitions dans ce domaine-

En novembre dernier, les pays membres de l'Agence spatiale européenne sont allés au-delà des espérances de cette agence, en lui accordant plus de 14 milliards d'euros sur trois ans, ce qui permettra de poursuivre les programmes historiques concernant l'exploration, les applications ou les lanceurs, mais aussi de développer de nouveaux programmes, pour répondre aux nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés, par exemple en matière de sûreté et de sécurité de l'espace. La volonté de l'Union européenne d'accompagner cet élan est moins claire. la proposition budgétaire initiale de la Commission témoignait d'une véritable ambition spatiale, avec 16 milliards d'euros sur sept ans, une somme saluée sur toutes les travées. Toutefois, la dernière proposition du président du Conseil européen a réduit cette enveloppe prévisionnelle à 13,2 milliards d'euros. Ces derniers mois, le Sénat a affirmé, dans deux résolutions européennes, son attachement au niveau de financement initialement envisagé. Charles Michel réunit aujourd'hui les membres du Conseil européen pour tenter d'obtenir un accord- ce n'est pas gagné -sur le prochain cadre financier pluriannuel. Savez-vous, madame la ministre, ce qui en sortira ? Je ne le crois pas, mais je pose tout de même la question. Le Gouvernement a indiqué à plusieurs reprises soutenir un financement ambitieux, mais n'y a-t-il pas, chez certains de nos partenaires, la tentation de préférer financer le secteur spatial l'ESA, qui applique le principe du retour géographique ? Ce serait une logique court-termiste qui ne ferait à terme que des perdants. Je l'ai rappelé à nos collègues représentants des parlements nationaux pas plus tard que ce mardi, lors de la conférence interparlementaire sur la stabilité, la coopération économique et la gouvernance en Europe qui était organisée au Parlement européen : tout ce que nous n'accomplirons pas au niveau de l'Union européenne, c'est sur notre budget national que nous devrons le prendre en charge, mais à une échelle moins pertinente, et donc moins efficace. Qu'en est-il du budget de la recherche ? Auditionnée récemment par la commission des affaires européennes du Sénat, la secrétaire d'État aux affaires européennes a indiqué que le Gouvernement visait désormais une enveloppe dédiée au spatial à l'intérieur du programme Horizon Europe de 2,5 milliards d'euros, quand nous réclamions 4 Ce n'est pas satisfaisant, à l'heure où les modifications radicales des technologies de l'écosystème spatial s'accélèrent. Nous devons nous donner les moyens d'accompagner les start-up innovantes, mais aussi anticiper les futurs développements de Galileo, de Copernicus et d'Egnos. Enfin, je vous appelle, mes chers collègues, à mener, dans vos territoires, la bataille de l'opinion publique. Thomas Pesquet, qui repartira l'an prochain dans la station spatiale internationale, demeurera, certes, le meilleur ambassadeur de notre ambition spatiale.

À l'heure des batailles de chiffres, quand les intérêts nationaux menacent de primer sur l'intérêt commun, regardons plus haut : c'est peut-être là que se construira le futur de notre Terre commune. La parole

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires européennes, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de remercier la commission des affaires européennes pour l'organisation de ce débat. Les questions spatiales demeurent trop souvent éloignées des débats en séance publique, et cela est évidemment regrettable. Chacun comprend bien à quel point les enjeux spatiaux sont consubstantiels à la défense de notre souveraineté et à la construction de notre prospérité économique, et je sais à quel point les commissions des affaires économiques, des affaires étrangères et de la défense et des affaires européennes sont engagées sur ces sujets. La question spatiale est au coeur des enjeux européens. Le séminaire Perspectives spatiales, que j'ai ouvert ce matin, le rappelle en ce moment même. Naturellement, cela est un acquis du traité de Lisbonne et de l'article 189 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui assignent à l'Union européenne l'obligation de se doter d'une politique spatiale en vue de favoriser le progrès scientifique et technologique, mais aussi de renforcer sa compétitivité industrielle. Cette politique fut historiquement- c'est toujours le cas aujourd'hui -le fruit d'une coopération renforcée entre les États de l'Union européenne. Les politiques spatiales des pays membres de l'Union contribuent ainsi à alimenter ses orientations propres dans le cadre proposé par l'Agence spatiale européenne. comme chacun le sait, joue un rôle leader dans la structuration de la politique spatiale de l'Union européenne. Nous le devons à des choix politiques forts et structurants qui garantissent à la France et à l'Union européenne d'appartenir au cercle des grandes puissances spatiales. Je songe également au rôle stratégique que jouent la Guyane et le centre de Kourou, qui, ainsi que le relève le rapport de votre commission des affaires européennes, est le véritable « port spatial de l'Europe », garantissant le libre accès de l'Union européenne à l'espace. Ce mode de fonctionnement, qui est le produit tant de l'histoire que de l'originalité même du projet européen, distingue d'emblée la politique européenne de celles des autres puissances spatiales, dont la politique est d'abord structurée autour des questions de défense. Cette originalité, si elle n'a jamais fait obstacle au succès de la politique européenne en matière spatiale, doit être questionnée à la lumière des enjeux actuels relatifs à la nouvelle donne qui s'impose dans la compétition spatiale. La politique spatiale de l'Union européenne n'a pas à rougir de la concurrence internationale. Le volume d'investissement annuel cumulé de l'Europe en la matière est tout à fait comparable aux investissements réalisés par la Chine. Au-delà des seules grandes masses financières, l'Union européenne peut revendiquer de réels succès. Je songe évidemment à Galileo ou à Copernicus, deux programmes qui témoignent par eux-mêmes de la spécificité de notre politique spatiale et de sa pertinence stratégique. La collecte de données et d'informations depuis l'espace représentera, dans les prochaines décennies, un enjeu majeur de développement économique et de prévention des risques en Europe et dans le monde. C'est l'un des enjeux du programme Copernicus. De même, en matière de transport et de géolocalisation, les applications de Galileo sont reconnues pour leur valeur ajoutée en comparaison du GPS ou des systèmes russes ou chinois. Galileo dépasse les frontières de la seule Union européenne et profite aujourd'hui à plus de 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Pour autant, si l'Europe dispose d'atouts indéniables, si elle est déjà riche d'un bilan remarquable en la matière, nous devons regarder avec lucidité la nouvelle donne à l'oeuvre dans le monde. Une course mondiale aux lanceurs est en cours, révélant une compétition pour l'accès le plus efficient à l'espace. La concurrence s'accroît, notamment du fait de la montée en puissance du secteur spatial asiatique ; je songe aux fusées Longue Marche chinoises ou aux fusées SLV indiennes. Bien que la mission Chandrayaan-2 ait échoué, l'Inde a clairement affirmé son intention d'envoyer des hommes sur la Lune, un objectif toujours partagé également par les États-Unis et la Chine. Au-delà des seules puissances étatiques, les dernières années ont vu l'émergence d'acteurs industriels puissants. Je songe naturellement au secteur du et à son porte-étendard, SpaceX, qui dispose à la fois d'une force de frappe inédite en matière de communication et qui poursuit surtout des objectifs ambitieux. Le groupe pourrait en effet bientôt disposer d'une constellation de 180 satellites tout en ayant annoncé son souhait de déployer plus de 40 000 appareils autour de la Terre. Cet investissement de l'espace n'échappe pas non plus aux GAFA. Blue Origin est ainsi une société dirigée par Jeff Bezos, le président-directeur général du groupe Amazon. Dans ce contexte, l'Europe doit tenir son rang et affirmer sa position de leader. Nous sommes confiants dans notre capacité à conserver ce rôle, à condition que nous continuions d'avancer dans un même mouvement au sein de l'Union européenne. Les engagements souscrits à Séville dans le cadre de l'ESA ont atteint 14,4 milliards d'euros, une somme supérieure à ce qui était attendu par l'Agence et représente une augmentation de 4 milliards d'euros par rapport à la précédente conférence ministérielle, témoignant d'une grande confiance collective dans le spatial européen. Ces engagements permettront d'impulser des projets ambitieux comme de garantir l'achèvement des programmes Ariane 6 et Vega C. En matière scientifique, la mission LISA nous permettra de progresser dans la détection des ondes gravitationnelles

la mission qui permettra le retour des échantillons de roches martiennes, le, pour disposer d'une station à mi-chemin entre la Terre et la Lune, ou encore le prochain retour en vol de Thomas Pesquet sur la station spatiale internationale. Naturellement, la France a joué un rôle déterminant dans le succès et l'ambition de la conférence de Séville, que j'avais l'honneur de coprésider. La souscription totale de notre pays a été de 2,7 milliards d'euros, des nouveaux engagements qui s'ajoutent à notre contribution annuelle

Au-delà des chiffres et des engagements financiers, il va de soi que, une politique spatiale, c'est aussi un récit sur l'aventure collective vécue par celles et ceux, dans vos territoires, qui dédient leur carrière et leurs rêves au secteur spatial. C'est un désir d'exploration et d'aventure, c'est un besoin de connaissance. Ce récit existe en Europe, et mon engagement en tant que ministre, c'est de travailler à le diffuser à une époque où la défiance envers le progrès scientifique et technologique se répand dans le débat public. Faire connaître ce récit, faire connaître cette politique, rappeler ce qu'elle apporte au quotidien à nos concitoyens, mais également à vos territoires, en termes d'activité et de développement économique, tout cela fait partie des enjeux de ce débat. Je tâcherai naturellement de répondre à l'ensemble de vos questions. Nous allons

parole est à M. Jean-Claude Requier. Vous avez bien présenté les perspectives de l'Union européenne en matière de politique spatiale et les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que Français et Européens. Il s'agit d'un sujet à la fois passionnant et essentiel, qui peut être un puissant levier de mobilisation des énergies et d'adhésion populaire. L'Europe a raison de s'en saisir, comme elle l'a annoncé il y a quelques mois, pour des raisons stratégiques. Ce que l'on comprend à la lumière du rapport de la commission des affaires européennes, c'est que le spatial devient de plus en plus un enjeu de souveraineté pour les Européens. La France reste une puissance spatiale qui compte, avec un budget de la recherche et un budget du CNES (Centre national d'études spatiales) parmi les grands budgets mondiaux ; grâce aussi, rappelons-le, au site de lancement de Kourou, en Guyane, qui fait de notre pays le seul État européen à disposer d'une capacité de lancement autonome. Le niveau européen n'est pas en reste, puisque le budget de l'Agence spatiale européenne est l'un des premiers au

Quelle est l'action de l'Union européenne et du Gouvernement français dans ce cadre ?

avec l'arrivée du, c'est-à-dire des nouveaux acteurs que vous avez cités, madame la ministre, tels SpaceX, qui cassent les prix de l'accès à l'espace, le spatial européen va au-devant d'une crise profonde. nous pouvons toujours nous féliciter des réalisations remarquables de l'Europe en matière spatiale, Galileo et Copernicus en tête ; elles sont indéniables, mais, si nous ne réagissons pas, elles pourraient bien s'apparenter au chant du cygne. Face à l'émergence du nouveau modèle spatial américain, la politique spatiale européenne doit se réinventer, économiquement mais aussi institutionnellement. De fait, le cadre institutionnel actuel, qui a permis au spatial européen de devenir l'un des meilleurs du monde, est aujourd'hui obsolète. Depuis le traité de Lisbonne, de 2009, l'espace est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres. Mais c'est l'Agence spatiale européenne, l'ESA, créée en 1975, qui est l'opérateur central du spatial européen. Or cette organisation internationale intergouvernementale repose sur le principe de l'unanimité. De plus, l'ESA est fondée sur la règle du retour géographique, en vertu de laquelle toute somme investie par un État membre dans un projet de l'Agence est dépensée dans l'industrie spatiale de ce pays : 1 euro investi rapporte 1 euro. Ce fonctionnement est totalement contraire aux principes de l'Union européenne Madame la ministre, étant donné que c'est le maintien de notre autonomie d'accès à l'espace qui est en jeu, n'est-il pas temps de procéder à un big-bang institutionnel consistant à basculer la gouvernance du spatial européen de la coopération vers l'intégration ? N'est-il pas temps que l'Union européenne Mme la ministre. la prédominance qu'avaient la France et l'Union européenne dans le domaine des lanceurs est aujourd'hui mise au défi par d'autres compétiteurs que ceux auxquels nous étions habitués. Évidemment, nous ne sommes

la guerre se déporte de plus en plus vers l'espace, dans l'espace lui-même mais aussi au sol, compte tenu de la dépendance de plus en plus grande des systèmes économiques et des troupes militaires à la géolocalisation.

allons-nous laisser perdurer la réticence du Japon, des États-Unis et de l'Europe à discuter d'un nouvel accord international protégeant l'espace ? Le américain de 2015, marquant une rupture unilatérale du traité de 1967, a autorisé les entreprises états-uniennes à s'emparer des ressources spatiales. Aujourd'hui, des acteurs privés majeurs sont subventionnés par le Pentagone, qui y consacre beaucoup d'argent. Pendant ce temps, nous prenons du retard, avec l'assèchement progressif d'ArianeGroup

Madame la ministre, il n'y avait aucune naïveté dans ma question. Je pense que, si nous nous laissons aspirer vers la militarisation croissante de l'espace en la considérant comme inéluctable, elle mangera les ressources que nous devons consacrer,

vient de l'évoquer. En effet, voilà des décennies que nous lançons fusées, satellites et autres engins qui restent en orbite, basse ou géostationnaire, autour de la Terre. Si bien que, désormais, on peut parler de déchets spatiaux et de pollution spatiale. Alors que l'Union européenne s'est dotée d'un paquet législatif pour donner de la circularité à son économie, elle devra, tôt ou tard, se pencher sur l'écocircularité des déchets qui gravitent à des milliers de kilomètres

Terre- sans parler des plus gros débris. Les conséquences peuvent être catastrophiques pour l'observation spatiale, mais aussi pour la navigation de nos satellites et fusées. Dans les

Dans ce contexte, madame la ministre, quel est l'engagement de la France au plan européen, compte tenu de son expérience dans la lutte contre la pollution spatiale ? Le futur programme spatial européen prendra-t-il en compte la limitation et le traitement des débris spatiaux ?

commencions tout de suite à penser à cette pollution par les débris spatiaux de notre environnement proche.

Dans sa résolution du 9 août dernier sur la politique spatiale de l'Union européenne, le Sénat a souligné la nécessité pour l'Union européenne de continuer à disposer d'un accès souverain à l'espace. Le général de Gaulle, le 21 mars 1964, a déclaré à Cayenne : « Nous avons à réaliser, vous, sur place, et la France avec vous, une grande oeuvre française en Guyane. »

au vu du contexte concurrentiel mondial : il doit impérativement se moderniser et remettre à niveau ses radars et stations de réception pour faire d'Ariane 6, dont le premier vol est prévu pour cette un lanceur durablement compétitif, notamment face aux progrès de SpaceX. Il lui faut également préparer la transition vers le réutilisable. L'accès L'accès souverain de l'Union européenne à l'espace suppose de mettre en place une préférence européenne dans le domaine des lanceurs, afin de soutenir les entreprises qui opèrent dans ce secteur. À l'issue du sommet de Toulouse, le 16 octobre dernier, la Chancelière Merkel et le Président Macron ont réaffirmé leur soutien au principe de préférence européenne en ce qui concerne les lanceurs, en particulier pour Ariane 6. Ce ralliement de l'Allemagne semble aplanir les dernières difficultés. Si je suis un élu guyanais soucieux des retombées du spatial pour mon territoire, je reste conscient que celles-ci reposent nécessairement sur la capacité du CSG à demeurer compétitif. Madame la ministre, peut-on Madame la ministre, peut-on désormais compter avec certitude sur la perspective d'une préférence européenne pour les lanceurs, susceptible de renforcer la compétitivité du Centre spatial guyanais et de consolider notre industrie spatiale ? La parole

depuis le début de l'ère spatiale, nous en avons envoyé 8 000. C'est dire sur quelle trajectoire- sans faire de jeu de mots -s'engage la colonisation de l'espace. Indépendamment de la question fondamentale de la pertinence, du besoin réel, des usages que ces satellites permettront sur notre Terre- peut, il devrait, y avoir débat là-dessus -, on ne peut s'empêcher de faire le parallèle entre la dégradation de l'écoumène terrestre et la pollution promise, si ce n'est déjà effective, de l'espace satellitaire. l'espace satellitaire. Il s'agit aujourd'hui d'un espace international peu régulé, et les sujets de préoccupation, si ce n'est d'inquiétude, sont multiples : d'abord, pour la gestion et le pilotage des engins, qui se sont complexifiés depuis l'arrivée en force des acteurs privés ensuite, pour la préservation de l'espace lui-même contre les débris et les pollutions diverses qu'engendre cette activité en forte croissance. Pour les orbites basses, inférieures à 600 kilomètres, le nettoyage se fait à peu près naturellement,

quelle est, s'il y en a une, l'ambition juridique internationale du Gouvernement pour que la France contribue, dans un contexte insuffisamment régulé, à préserver l'espace de toute pollution d'origine terrestre ?

Vous avez raison, il n'existe pas, à ce jour, de traité international garantissant l'effectivité de cette désorbitation. C'est pourquoi, là aussi, il est très important

par les opérateurs de satellites est le standard ISO 24113, qui n'est pas opposable juridiquement. Cette norme a pour objectif d'empêcher la création de nouveaux débris dans l'espace.

Aujourd'hui, il existe trois piliers. Premier pilier : l'Union européenne, avec la nouvelle direction générale défense et espace, Copernicus et Galileo. Deuxième pilier : l'ESA, l'Agence spatiale européenne, à laquelle participent également des pays non membres de l'Union européenne, comme, depuis le Brexit, le Royaume-Uni, mais également la Norvège, la Suisse et des pays associés tels que le Canada. Troisième pilier : les agences nationales, c'est-à-dire, en France, le CNES mais encore la DGA et le nouveau commandement de l'espace, placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air. On voit donc bien que, au travers de tous ces piliers, il y a un manque de synergie, de coordination. Certes, il existe le conseil Espace, qui veille à rapprocher l'ESA de l'Union européenne, mais cela n'est pas suffisant. Je vais prendre deux exemples pour illustrer mon propos. Premier exemple : l'exploitation minière de la Lune, décidée par les États-Unis et à laquelle s'associe le Luxembourg,

en matière spatiale ; j'y participe de manière évidemment très régulière. L'implication de la France dans le budget de l'ESA représente 2,7 milliards sur un budget de 14,4 milliards d'euros pour les trois années à venir ; c'est une contribution importante, qui s'ajoute, je l'indiquais, aux contributions annuelles de la France.

partagez-vous cette inquiétude et cette urgence ? Au-delà de Prometheus et d'ArianeWorks, quelle est la logique du rapport de force entre lanceur satellitaire et utilisateurs de l'espace ? La parole est

En termes de compétitivité, nos entreprises ont réalisé un énorme travail entre Ariane 5 et Ariane 6, puisque Ariane 6 sera 40 % moins chère qu'Ariane 5, tout en gardant la capacité à atteindre absolument toutes les orbites et à pouvoir embarquer des satellites beaucoup plus importants.

pour la réplique. Madame la ministre, je vous suggérerais que le Gouvernement français saisisse l'OMC de la déloyauté des prestations de SpaceX

pression susceptible de remettre en cause notre indépendance dans l'accès à l'espace. Cette très forte pression provient, nous le savons, des concurrents américains, dont SpaceX, qui bénéficient de commandes institutionnelles fort bien payées et qui ont développé la seule rupture technologique réussie réussie dans le domaine des lanceurs depuis le lancement de Spoutnik en 1957 : la réutilisation du premier étage. Par ailleurs, tous les gouvernements européens ne sont pas également convaincus de la nécessité de maintenir un accès autonome à l'espace, ce qui rend certains réticents à contribuer mieux et plus avant au programme de développement des lanceurs. Dans ce contexte, la dernière chose dont l'Europe a besoin est d'une concurrence fratricide. C'est pourquoi nous avions alerté, avant la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, sur la nécessité d'être extrêmement prudents sur le programme Vega E, proposé par l'Italie Vega est une grande réussite,

compétition potentielle fait l'objet de discussions permanentes, à la fois avec le gouvernement italien, mais aussi entre les industriels. Toutefois, n'oublions pas que Vega et Ariane

a dû être dévié de sa trajectoire pour éviter une collision avec l'un des satellites de Starlink 44. Ma question est très simple : ne risque-t-il pas, à terme, de ne plus y avoir d'espace dans l'espace ?

Les lanceurs Ariane 4 et 5 en sont l'expression la plus achevée. Les entreprises européennes ont aussi conçu des satellites de très grande qualité et très performants. Cette politique, soutenue continûment par les États partenaires, nous a permis d'être indépendants, tant dans le domaine civil que sur

à des retards de lancement. Un autre, et non des moindres, est que chaque lancement coûte très cher en subventions aux États, donc aux contribuables. La concurrence est vive dans le domaine commercial. le domaine commercial. SpaceX a de plus en plus de succès. Il fallait donc réagir. Le programme Ariane 6 a été conçu et décidé en 2014 et développé par ArianeGroup. Ce lanceur plus petit pourra n'emporter qu'un seul satellite, ce qui lui donnera plus de souplesse, et le dernier étage sera réallumable, ce qui lui offrira plus de plus de possibilités en cas d'emport de plusieurs satellites dont les orbites sont différentes. Le premier lancement est prévu pour juillet 2020. Au vu de ces enjeux, madame la ministre, la réorganisation de la filière spatiale et les choix techniques retenus pour Ariane 6 permettront-ils de réaliser des lancements économiquement compétitifs par rapport à ceux que propose SpaceX ? Des subventions sont-elles encore nécessaires pour équilibrer le budget ?

Oui, nous avons toujours besoin d'accompagner la filière spatiale, pour la simple raison que nous devons accompagner la transition entre Ariane 5 et Ariane 6. Chaque fois qu'un nouveau lanceur est mis sur le marché, il y a une hésitation et donc une baisse

Le fait est que SpaceX, largement soutenu par la NASA, maîtrise la récupération et la réutilisation du premier étage, ce qui est préjudiciable à la compétitivité de notre lanceur par rapport à celui des Américains.

Avec l'émergence de nouveaux acteurs étatiques et privés, la dernière décennie a été le théâtre d'une transformation rapide et profonde de l'économie du secteur spatial. La concurrence exacerbée qui s'exerce désormais sur ces marchés de plus en plus stratégiques a érodé la position des industriels européens, qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de l'ordre de 3 % en 2018. Le secteur des lancements, qui commande ni plus ni moins que l'accès à l'espace lui-même, est bien évidemment particulièrement touché. En 2019, l'Europe s'est fait largement distancer, au nombre de tirs réalisés, par la Chine, les États-Unis et la Russie. L'une des raisons de cette perte de vitesse réside, à mon sens, dans le volume trop faible de la commande publique. En effet, là où le carnet de commandes de SpaceX

Dans ce contexte, il est nécessaire de consentir aux efforts budgétaires à même d'accroître la commande publique et de mieux structurer le marché institutionnel, mais il est également indispensable de progresser plus rapidement et de manière plus affirmée sur la voie de la préférence européenne, qui a plusieurs fois été évoquée dans ce débat. Nos concurrents n'ont aucun état d'âme à imposer une telle préférence nationale pour leur lancement satellitaire. Nous n'y sommes

-du règlement pour le programme spatial européen. Toutefois, il manque encore l'outil clair et contraignant garantissant l'engagement de tous les donneurs d'ordre publics.

le passage d'Ariane 5 à Ariane 6 a nécessité de repenser jusqu'au pas de tir du lanceur, nous travaillons avec les industriels

La question de la préférence européenne a été au coeur des discussions de ces deux dernières années. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, maintenant que le Bundestag a voté en ce sens, plus rien n'empêche cette préférence européenne. Nous en parlerons lors du prochain conseil, mais je pense que c'est désormais acté, du moins du point de vue des plus gros lanceurs.

de la culture pour les crédits de la recherche, j'observe avec satisfaction que les vingt-deux États membres de l'Agence spatiale européenne ont souscrit plus de 14 milliards d'euros de programmes pour les trois à cinq prochaines années lors du conseil ministériel de l'ESA qui s'est tenu à la fin du mois de novembre dernier à Séville. De la même façon, nous pouvons nous réjouir que la Commission européenne ait prévu d'inscrire 16 milliards d'euros de crédits pour la période 2021-2027 au profit des deux programmes majeurs que sont Galileo et Copernicus et de deux programmes plus récents, consacrés l'un aux satellites gouvernementaux, l'autre à la surveillance des objets en orbite. Permettez-moi, à cet instant, de saluer l'action continue du président du CNES, Jean-Yves Le Gall, qui permet à la France, mais aussi à l'Europe, d'être toujours dans la course spatiale mondiale. Toutefois, les défis à relever sont immenses. Le secteur spatial français et européen est confronté à une forte concurrence internationale celle des États, d'une part, avec le renforcement de puissances émergentes comme le Japon, la Chine et l'Inde, et l'apparition de nouveaux acteurs, à l'image des Émirats arabes unis ; celle des acteurs privés, d'autre part, avec les sociétés SpaceX, présidée par Elon Musk, et Blue Origin, dont le président n'est autre que Jeff Bezos, le président d'Amazon, qui investissent lourdement dans le secteur spatial.

Mme la ministre.

qui témoignent non seulement d'un vif intérêt pour le sujet de l'espace, mais aussi d'une connaissance approfondie des enjeux de ce secteur, tant techniques et économiques que géopolitiques et sociétaux. Ayant demandé l'inscription de ce débat à l'ordre du jour au nom de la commission des affaires européennes, j'insisterai, en conclusion, sur la sur la valeur ajoutée de l'échelon européen pour affronter les enjeux du secteur spatial. Dans cette perspective, je reviendrai sur deux points. D'abord, c'est dans ses applications que se trouve désormais la valeur ajoutée de l'écosystème spatial, avec plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année, contre environ 6 milliards d'euros, par exemple, pour les lanceurs. C'est là aussi que se trouvent les plus grands relais de croissance. L'Union européenne devra donc jouer un rôle majeur, dans les mois et les années à venir, pour maximiser les retombées à la fois économiques

La Commission européenne a présenté hier sa stratégie pour les données, mentionnant notamment un européen souverain, un accès centralisé aux données et aux outils de traitement. Cela existe d'ailleurs déjà en partie pour Copernicus, avec les plateformes DIAS. Nous suivrons attentivement la mise en oeuvre de ce plan. Par ailleurs, un accès souverain à l'espace est une nécessité stratégique pour l'Europe. Le Sénat réclamait déjà, dans sa résolution européenne du 9 août dernier, que l'Union fasse preuve de volontarisme dans son soutien aux lanceurs spatiaux européens et mette en place une préférence européenne au bénéfice de ses entreprises qui opèrent dans ce secteur : une préférence de droit, mais aussi de fait,

en orbite des satellites Galileo. Je souhaite que la dynamique se poursuive, voire puisse s'amplifier. Il faudrait aussi réfléchir à la possibilité d'une préférence européenne pour les commandes institutionnelles de satellites. L'aventure spatiale fait rêver, mais gardons-nous de tout angélisme. Des actions convergentes se mettent en place pour donner à l'Europe les moyens d'une ambition spatiale. Cette ambition est une nécessité